L’amitié, comme l’amour, demande beaucoup d’efforts, d’attention, de constance, elle exige surtout de savoir offrir ce que l’on a de plus cher dans la vie : du temps

aux élus et faire en sorte que le temps d’absence légale d’un élu soit considéré comme du temps de travail effectif.

En effet, un salarié qui souhaite s’engager dans la démocratie locale ne doit pas être pénalisé. Le temps qu’il consacre à sa mission d’élu est d’une grande richesse pour la collectivité. Par cet amendement, nous vous invitons donc à faire en sorte que le temps d’absence légale d’un élu soit considéré comme du temps de travail

En application de ce principe, lorsque ce temps d’absence n’est pas rémunéré par l’employeur, l’assiette des cotisations ne doit pas s’en trouver réduite. Ce principe nécessite cependant d’être mieux connu, car il n’est pas toujours respecté. Tel est l’objet

à du temps de travail effectif pour le calcul du bénéfice de certains avantages sociaux, sans remettre en cause l’absence d’obligation pour l’employeur de rémunérer ce temps. Les élus locaux bénéficient d’autorisations d’absence pour participer aux réunions inhérentes à leurs fonctions. Elles sont accordées aux membres du conseil municipal, départemental et régional.

Le fait de viser les droits liés à l’ancienneté a justement pour objectif de garantir au salarié élu le maintien de tous ses droits en matière de salaire : primes, titres restaurant et autres accessoires de salaire. Vos demandes sont donc déjà satisfaites, mesdames, messieurs La modification du régime du congé de représentation que vous proposez à cet effet est non seulement inutile, mais inadaptée. À l’inverse, supprimer la formulation relative au droit à congés payés et aux droits liés à l’ancienneté rendrait le droit moins lisible, particulièrement en matière de durée du temps de travail et de contrôle des durées maximales du travail. Le respect des durées maximales de travail repose sur les entreprises ; or, en assimilant le temps d’absence légale à du temps de travail, les entreprises risquent de ne plus avoir de contrôle sur les durées maximales de travail. De plus, le droit en vigueur prévoit déjà des protections importantes. Les garanties accordées aux élus sont déjà considérables pour l’employeur, qui est contraint de prendre en compte le statut d’élu local de ses employés dans l’organisation et le fonctionnement de son entreprise.

le statut de salarié protégé pour les maires et adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants. Il nous semble qu’il est grand temps de le rétablir et de l’étendre à l’ensemble des élus locaux. Par cet amendement, nous nous engageons à protéger les élus locaux au même titre que les représentants syndicaux. Cette protection est la garantie de l’indépendance des élus : elle permet de leur donner les moyens de s’engager et d’œuvrer pour l’intérêt général. proposons que le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne puisse intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. Mes chers collègues, cet amendement

les élus locaux ont déjà bénéficié de cette protection. Malheureusement, comme l’avait noté la délégation aux collectivités territoriales en 2018, ce statut était inapplicable, faute de dispositions inscrites dans le code du travail. Plutôt que de corriger cette anomalie, la loi Engagement et proximité a supprimé

Les indemnités de fonction, la plupart du temps très modestes, ne peuvent en effet constituer un revenu de remplacement. Or, si des dispositions légales existent pour permettre aux élus locaux ayant conservé une activité salariée de disposer du temps nécessaire pour l’exercice de leur mandat je pense notamment aux crédits d’heures trimestriels et aux autorisations d’absence –, la protection qu’offre le code du travail leur fait actuellement défaut. C’est pourquoi je propose, avec cet amendement, de placer les élus locaux salariés,

présente proposition de loi encourage la mise en place de mécanismes incitant les entreprises à se mobiliser en faveur des élus. Toutefois, nous pensons qu’il est possible d’aller plus loin, en étendant à ces élus des dispositifs existant pour les salariés protégés.

d’autre part, des communes de plus de 10 000 habitants étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail

de salarié protégé vise à assurer l’effectivité de la démocratie sociale, du droit syndical et du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises.

: il permet de garantir aux représentants du personnel l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur mandat et de les protéger contre les mesures arbitraires auxquelles leurs fonctions les exposent.

Une telle protection avait été instituée dans le code général des collectivités territoriales par la loi n° 2015 366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat,

Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. En effet, En effet, constatant que la reconnaissance d’un statut de salarié protégé aux élus ne leur assurait pas une protection effective, et que, par ailleurs, elle pouvait contribuer à dissuader les employeurs d’embaucher des candidats titulaires de mandats locaux

qui ont besoin que la puissance publique leur vienne en aide. Je suis d’accord avec vous, madame la ministre, il ne s’agit pas de confondre l’engagement syndical et l’engagement politique. Pour autant, nous devons veiller à la défense des corps intermédiaires,

qui nous a expliqué par le menu ce qu’il a dû affronter pour pouvoir exercer convenablement son mandat d’élu, et tous les obstacles, pour ne pas dire pire, qu’il a dû surmonter. Cela justifie pleinement que nous

je vous rappelle que

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

de la présente proposition de loi appellent deux réflexions. En premier lieu, il me paraît essentiel de laisser l’entreprise faire ce qu’elle sait faire de mieux, à savoir produire et créer de la valeur.

Au prétexte d’un État qui ne voudrait pas assumer la démocratie locale comme précepte fondateur de la République, ne nous laissons pas dériver dans des eaux troubles, vers un mélange des genres qui tuerait, à terme, notre démocratie de proximité. chers collègues, la crise de la démocratie est profonde. N’en ajoutons pas et n’exposons pas les élus locaux à des risques de conflits d’intérêts ; ne jetons pas en pâture ceux qui bénéficient encore de la confiance des Français

Miquelon. Quel est l’avis de la commission ?

d’évoquer avec leur employeur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et exercice du mandat et de valoriser les compétences acquises à l’issue de celui ci. Le présent amendement vise à étendre cette mesure aux fonctionnaires titulaires d’un mandat local. Quel est l’avis de la commission

pour se rendre aux séances et réunions donnant droit à des autorisations d’absence pour les élus salariés. Le Gouvernement est très favorable à une extension des modalités de remboursement des frais de déplacement pour l’ensemble des élus. C’est pourquoi nous vous proposons d’assouplir les dispositifs prévus à cet effet dans le code général des collectivités territoriales,

13 comporte des avancées significatives : une aide financière à la préparation des réunions, le relèvement du plafond de prise en charge des avances de frais, une prise en charge directe par la commune des aménagements des postes de travail.

mais qu’il remette un rapport étudiant sérieusement la question de la mise en place d’une structure nationale de compensation du handicap pour les élus, dotée d’un fonds dédié pour une prise en charge complète, personnalisée et sans avance

malgré de multiples sollicitations. J’ai personnellement saisi cinq fois les ministres successifs chargés des personnes en situation de handicap, par courrier et par question écrite. Quand j’ai obtenu une réponse, celle ci était incomplète

à une élection locale. L’article 14 crée ainsi un nouvel article L. 325 8 1 dans le code général de la fonction publique qui prévoit que chaque statut particulier fixe les conditions dans lesquelles les épreuves du troisième concours assurent la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant d’une activité professionnelle,

du II du présent article, qui s’appuie sur une définition du « candidat déclaré publiquement », laquelle n’est pas sûre juridiquement. En outre, la possibilité pour le candidat de financer une formation élective grâce à son compte personnel de formation

une formation, obligatoire mais nécessaire, à la compréhension des enjeux et des conséquences de ces violences pour l’ensemble des élus locaux. Dans le cadre de leur mandat, ces derniers doivent connaître le cadre juridique, savoir détecter, se positionner et réagir de la bonne manière face aux situations de VSS, et plus largement,

est l’avis de la commission sur les trois amendements

Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Le scrutin est clos.

Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

votre amendement vise à prévoir que le tribunal de grande instance organise, dans les trois mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, une réunion avec les maires de son ressort pour leur exposer le périmètre de l’exercice de leur pouvoir de police. Tribunal de grande instance » et « exercice du pouvoir de police » ? Oui, cela ne va pas… Non, en effet. Si le renforcement du dialogue institutionnel entre les parquets et les élus locaux figure au rang des priorités du ministère de la justice,

une autorité de police administrative et possède à ce titre des pouvoirs de police générale et spéciale lui permettant de mener des missions de sécurité et de tranquillité publique, il exerce ces pouvoirs sous le contrôle du juge administratif et non pas du tribunal judiciaire.

est l’avis du Gouvernement ? L’objet du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou à des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatifs sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

au maintien total par l’employeur de sa rémunération. Ce dernier verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. Le fait que l’entreprise rémunère ce congé pour des salariés exerçant un mandat d’élu local nous paraît d’élu local nous paraît disproportionné. De manière générale, les garanties accordées par le code du travail aux salariés élus – je les ai rappelées précédemment – correspondent à un équilibre satisfaisant entre l’exercice d’un engagement politique du salarié, que nous voulons encourager fortement, les contraintes assujetties à l’entreprise et les impératifs liés au bon fonctionnement

L’augmentation de l’indemnité des élus viendra mécaniquement renforcer le budget du Dife. Ainsi, les dispositifs de reconversion professionnelle, notamment les bilans de compétences, pourront bénéficier de financements qui permettront à ces élues de ne pas engager leurs deniers personnels

Cette session de deux jours, à suivre dans les trois premiers mois de mandat, est conçue pour approfondir leur compréhension des responsabilités, des droits et des obligations, notamment déontologiques, liés à leur fonction. L’objectif est d’assurer une prise de fonction éclairée et responsable, contribuant ainsi à une gouvernance locale plus informée et efficace.

relation avec les étrangers, y compris nos voisins européens, relève de votre responsabilité. Faites pression sur votre préfet pour qu’il inscrive ce point à l’ordre du jour d’une prochaine conférence intergouvernementale

Dans cette perspective, il étend aux communes de moins de 10 000 habitants la compensation par l’État des frais de garde engagés par les élus pour la participation aux réunions liées à l’exercice de leur mandat. Il crée également un nouveau dispositif pour les seuls exécutifs municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, leur ouvrant droit à la prise en charge des frais de garde pour leur participation aux activités liées à l’exercice de leur mandat. En accord avec le Gouvernement, nous proposons d’étendre cette compensation afin de l’harmoniser avec celle qui est prévue pour les coûts liés à la souscription d’un contrat d’assurance, au titre de la protection fonctionnelle des élus, qui a été élargie aux communes de moins de 10 000 habitants par la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cet amendement vise à compléter les dispositifs existants pour l’ensemble des élus, et non les seuls exécutifs des communes de moins de 3 500 habitants.

à la souscription d’un contrat d’assurance au titre de la protection fonctionnelle des élus, qui a été élargie aux communes de moins de 10 000 habitants par la loi de finances pour 2024 ; chacun l’a bien en tête. Si le Gouvernement est également favorable au renforcement de la prise en charge des frais de garde, la création d’un dispositif plus avantageux bénéficiant aux seuls exécutifs des communes de moins de 3 500 habitants ne semble pas justifiable au regard des exigences

Monsieur Blanc,

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du chèque emploi service universel (Cesu) à l’ensemble des élus. Le code général des collectivités territoriales permet aux collectivités d’accorder, par délibération, une aide financière à leurs élus qui utilisent des Cesu pour régler leurs frais de garde et d’assistance. Cette aide, dont le montant maximal est fixé par décret, ne peut se cumuler avec le dispositif de prise en charge des frais de garde. Elle ne peut être versée qu’aux seuls élus

accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, de nombreuses mesures législatives ont été prises pour renforcer la lutte pour l’égalité des femmes et des hommes dans les instances politiques de nos collectivités locales.

Toutefois, si nous pouvons nous féliciter de cette nette amélioration, nous ne pouvons nous en satisfaire. Certes, la représentation des femmes dans les instances délibératives locales a progressé, mais l’accès à la représentation dans les instances intercommunales et dans les exécutifs locaux leur est toujours plus difficile que pour les hommes.

le second est encore ignoré par nos institutions. Pourtant, il est aussi néfaste que le premier, car il affecte la détermination des femmes à endosser des responsabilités politiques au sein de nos collectivités. Aussi est il impératif d’engager une réflexion globale et moins institutionnelle sur les freins à l’engagement des femmes,

Il est inspiré des droits des salariés du secteur privé, qui bénéficient d’un maintien de salaire pris en charge par leur employeur. Ces dispositions s’appliqueront en cas de congé paternité ou d’adoption, ce qui présentera également l’avantage de faciliter l’articulation et la répartition

de loi. Pleinement consciente de la nécessité de renforcer la couverture sociale des élus qui cessent d’exercer leur mandat dans les cas déjà prévus de maladie, de maternité, de paternité ou d’accident, je souhaite y ajouter les cas d’accueil d’enfant et d’adoption.

des collectivités territoriales permettent à la collectivité de maintenir le versement des indemnités de fonction d’un élu qui ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, de maternité, de paternité ou d’accident. Le montant de l’indemnité qui lui est versée est alors au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Actuellement, cette compensation ne peut pas être versée aux élus qui ont cessé d’exercer totalement leur activité professionnelle et ne concerne pas les cas de congé d’accueil de l’enfant et d’adoption. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle afin de couvrir l’ensemble des élus percevant une indemnité de fonction et à étendre le dispositif de compensation par la collectivité en cas de congé d’accueil

Sautarel. L’alinéa 2 de l’article 17 prévoit qu’un élu local placé en arrêt maladie peut poursuivre l’exercice de son mandat sauf indication contraire du médecin lui ayant prescrit ledit arrêt. Ce dispositif entraînerait une réécriture de l’article L. 323 6 du code de la sécurité sociale et inverserait le principe actuellement collègue Alexandra Borchio Fontimp propose de supprimer cet alinéa et de conserver la rédaction actuelle de l’article susvisé, disposant qu’un élu local placé en arrêt maladie peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par par le médecin. L’autorisation médicale préalable permet en effet de mieux garantir la préservation de la santé de l’élu concerné et le protège également de tout soupçon de fraude. Quel

L’autorisation effective du médecin prescripteur est en effet essentielle pour que l’assuré continue à exercer son mandat local pendant son arrêt de travail. Eh oui ! Le médecin est là pour déterminer si l’état de santé de l’élu est compatible ou non avec cet exercice. Et c’est grâce à ce contrôle protecteur que les élus locaux sont assurés de pouvoir déroger à la réglementation relative aux arrêts de travail en continuant à exercer leur mandat dans des conditions qui leur permettent de voir leur état de santé préservé tout en étant assurés de percevoir leurs indemnités journalières pour maladie versées par la sécurité sociale. Je vous remercie, monsieur le sénateur, de cet amendement. La parole est à Mme le rapporteur.

d’enfant. Les élus qui cotisent sur leurs indemnités de fonction ont bien droit aux indemnités journalières au titre de leur mandat sous réserve de remplir les conditions d’ouverture. Celles ci constituent des revenus de remplacement et ne compensent pas, dans sa totalité, la perte de rémunération de l’assuré. En outre, les élus locaux ne bénéficient pas de dispositifs de couverture complémentaire pris en charge par l’employeur, comme cela est le cas pour la majorité des salariés. prévoit néanmoins un mécanisme de compensation pour les élus qui perçoivent des indemnités de fonction et qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. La collectivité maintient ainsi le versement des indemnités de fonction d’un élu qui ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident. L’élu perçoit donc au plus la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités

elle ne pourra pas bénéficier d’une compensation pour la perte de ses revenus, suspendus pendant le temps de son congé maternité. La question qui se pose est donc simple. Les élus sont souvent amenés à cesser leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat, n’ayant pour seul revenu que les indemnités liées à leurs fonctions au sein de leur mairie, et se retrouvent souvent moins bien couverts que leurs homologues ayant poursuivi une activité professionnelle. Alors que seulement 20 % des maires sont des femmes, qu’elles représentent plus de 50 % de la population, nous souhaitons reconnaître, encourager et faciliter l’accès des femmes aux responsabilités locales. Le congé maternité

l’amendement n° 47 rectifié. La décennie 2020, marquée par la pandémie, a amorcé une profonde évolution du rapport au travail des individus, qui accordent une plus grande importance

Nous devons être en phase avec les attentes de ceux que nous représentons et accompagner ce mouvement de transformation majeure qui touche toutes les strates de notre société. que les actifs s’interrogent sur le sens de leur travail, les élus locaux, quant à eux, sont de plus en plus nombreux à douter du sens de leur engagement politique du fait de la dureté des conditions d’exercice de leur mandat, de leur sentiment d’abandon, de leur impression d’être laissés sans soutien en première ligne, de la remise en cause de la légitimité de la démocratie représentative et de la montée en puissance des violences verbales,

d’exercer leurs fonctions pour prendre le temps nécessaire pour accueillir un enfant dans le cadre d’un congé maternité, maternité ou d’adoption de continuer à percevoir leurs indemnités de fonction. Il s’agit tout simplement, comme c’est le cas pour bien d’autres salariés en France, de leur accorder des moyens suffisants pour jouir pleinement et sereinement de la période si particulière dans une vie familiale que représente l’arrivée d’un enfant. Ils sont bien souvent totalement dévoués à leurs concitoyens, vous ne le savez que trop bien, mes chers collègues, mais ce dévouement ne devrait pas les contraindre à renoncer à leur mandat pour des raisons personnelles. C’est la raison pour laquelle je vous encourage à voter pour cet amendement. La parole

Nous partons de l’idée que l’absence d’une obligation de casier vierge pour les candidats à des élections est source de blocage dans la confiance entre les citoyens et les élus. Comment expliquer à nos concitoyens qu’un élu n’a pas l’obligation de produire un casier judiciaire vierge alors que plus de 400 professions l’exigent Cet amendement nous offre l’occasion d’y remédier en ajoutant une nouvelle condition d’inéligibilité pour l’élection des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais, pour se porter candidat, si cet amendement était adopté, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

diffusion de tout enregistrement présentant un caractère sexuel, la proposition sexuelle à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique, l’acquisition, la détention et la diffusion d’images pédopornographiques. Nous souscrivons

Il n’est nullement question ici de remettre en cause l’obligation de transparence et de probité auxquelles nous sommes tous attachés. pour atteindre cet objectif, il est important que les règles soient claires et qu’elles n’aboutissent pas, par un effet de balancier ou par un excès de suspicion, à décourager

Ghislaine Senée. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à un assouplissement trop large de l’infraction de prise illégale d’intérêts. L’article 18 exclut les intérêts publics des intérêts susceptibles de constituer l’infraction, considérant que la responsabilité pénale d’un élu ne peut être engagée du fait de la défense d’un tel intérêt. Nous nous inquiétons de cette formulation trop large et trop vague, qui risque d’affaiblir juridiquement le délit de prise illégale d’intérêts. Une appréciation au cas par cas par le juge des intérêts publics comme privés de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance et l’objectivité de l’élu est

permettent de corriger deux anomalies. D’une part, les conseils régionaux et départementaux ne sont pas soumis explicitement aux principes selon lesquels une délibération est illégale lorsqu’un conseiller intéressé à l’affaire y prend part, alors que les règles en matière de prévention des conflits d’intérêts leur sont également applicables.

a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission. Au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes, cela est assez explicable. Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs non seulement dans une situation d’insécurité juridique dans laquelle tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionné, à la merci des candidats évincés vindicatifs. Cela les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralentit et renchérit fortement les procédures de passation des contrats publics. Aussi, il convient de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que celui ci est constitué seulement quand un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée – ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel – et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.

cet amendement proposent de restreindre le champ d’application du délit de favoritisme, afin de préciser que celui ci n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique. Ils reprochent à ce délit de réprimer tout manquement, même involontaire, au droit de la commande publique. Ces critiques ne sont pas justifiées. La caractérisation de ce délit exige un élément intentionnel. Il n’est pas utile de préciser que le manquement doit être délibéré pour pour caractériser le délit de favoritisme dans la mesure où, conformément à l’article 121 3 du code pénal, il n’y a « point de crime ou de délit sans intention de le commettre raison pour laquelle toute infraction pénale nécessite pour être constituée que soit rapportée la preuve d’un élément moral ou intentionnel. Par ailleurs, la caractérisation du délit de favoritisme exige déjà que la violation de la réglementation procure un avantage. Certains manquements, par exemple l’absence de mise en concurrence,

cette disposition est source d’insécurité juridique pour les superviseurs, qui pourraient l’interpréter notamment comme exigeant un contrôle accru des personnes politiquement exposées. Pour répondre à ce problème, identifié par les sénateurs, le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer dans la loi, de manière claire et explicite, le principe d’une approche par les risques. En effet, si la loi impose aux entités assujetties la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcées ou complémentaires vis à vis de leurs clients ou bénéficiaires effectifs qui sont identifiés comme personnes politiquement exposées, l’approche par les risques exige une modulation de l’intensité et de la fréquence de ces mesures en fonction de l’appréciation qu’elles font

189 rectifié. Autant vous dire que nous demandons la suppression de cet article ! Après le contrat d’engagement républicain pour les associations de la loi Séparatisme, après la tentative de demander aux migrants de jurer respect aux lois

là, c’est normal –, ainsi que « les lois et les symboles de la République », et qu’il « s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public ». Il dispose également que le maire ou le président de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités s’engage publiquement à respecter ce serment.

apportent concrètement. Ensuite, mes chers collègues, nous examinons ici un texte censé faciliter la vie des élus, lever les ambiguïtés, fluidifier le travail

les valeurs de la République. Ils les respectent tous les jours, ne serait ce qu’en s’engageant au quotidien pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Pourquoi les pointer ainsi du doigt ? J’aimerais bien que vous puissiez nous dire quel élu ou collectif d’élus locaux a bien pu demander l’inscription dans le texte d’un article aussi déconnecté des réalités du terrain. Enfin, cet article

est à Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Pierre Jean Rochette vise à soulager la charge administrative des élus locaux concernés par les obligations déclaratives de la HATVP, en prévoyant que les services de la Haute Autorité préremplissent les déclarations d’intérêts, à l’instar de ce qui se fait pour les déclarations de

est favorable à ce que les élus locaux puissent valoriser, dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience, les compétences acquises à l’occasion de l’exercice de leur mandat. Pour mémoire, les élus locaux sont d’ores et déjà éligibles aux actions de VAE, l’article L. 6111 1 du code du travail énonçant que toute personne est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ». Une réforme importante de la VAE a été portée par le Gouvernement et les premières mesures sont entrées en vigueur le 1 janvier 2024. Elles sont marquées par le souci de simplification et de raccourcissement des délais. Les I à IV du présent amendement visent à rendre cohérente la rédaction du dispositif juridique qui encadre la VAE, la formation professionnelle et l’accès au bilan de compétences pour les élus locaux avec le droit commun. La VAE est aujourd’hui accessible à toute personne dans les conditions prévues dans le livre IV de la sixième partie du code du travail, sans qu’il soit besoin de préciser que les élus municipaux, départementaux ou régionaux sont éligibles. éligibles. En outre, l’article 25 fixe des conditions moins favorables pour les élus locaux, puisqu’il prévoit de réunir le jury jusqu’à six mois après le dépôt du dossier de validation, alors que le droit commun prévoit désormais un délai maximal de trois mois pour la présentation du candidat devant le jury à compter du dépôt du dossier de validation.

peuvent d’ores et déjà faire reconnaître par le biais de la VAE les compétences acquises dans le cadre de leur mandat, d’autre part, que le dispositif de certification mis en place au bénéfice des représentants du personnel et des mandataires syndicaux repose sur l’existence de titres professionnels délivrés par le ministère du travail.

il vise à confier au seul ministre chargé des collectivités territoriales la tâche d’établir la certification professionnelle

souvent difficile et délicat, le départ n’étant de plus pas toujours souhaité. Cette proposition de loi prévoit un certain nombre de dispositions pour accompagner les élus dans leur vie après

d’au moins un mandat pourraient être admis en deuxième année d’une formation universitaire de droit, de sciences politiques, d’économie ou d’administration. Quel

ayant exercé deux mandats la voie de promotion interne créée par la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, à savoir la nomination dans un cadre d’emploi de catégorie B, en l’espèce de rédacteur territorial, après examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante. Cette proposition n’est pas sans poser des difficultés, qu’il s’agisse de la possibilité pour un ancien élu d’être recruté dans la collectivité dont il aurait été l’élu ou du financement du suivi de la formation qualifiante par cet élu. Tout d’abord, il ne paraît pas envisageable que la collectivité finance la formation d’un élu sur les crédits de formation de son personnel ni que le Centre national de la fonction publique territoriale la prenne en charge. De ce fait, l’adoption de l’amendement créerait une charge nouvelle, ce qui semble irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution. Surtout, une voie de promotion interne ne peut être ouverte qu’aux seuls agents publics. L’élu local n’est pas un agent public au sens du code général de la fonction publique et ne peut donc bénéficier de ce dispositif, à avoir la qualité de fonctionnaire indépendamment de son mandat. Les élus locaux disposent d’ores et déjà d’un accès à la formation publique par la voie du troisième concours, ainsi que le rappelle l’article 14 de la proposition de loi. Pour ces raisons, j’émets donc un avis défavorable

ces listes d’aptitude sont réservées aux agents publics, les agents étant présentés par les communes. Je ne vois pas comment le président ou la présidente d’un centre de gestion peut recevoir des dossiers indépendamment de cette trajectoire.

et des établissements publics de coopération intercommunale, géré par ailleurs par la Caisse des dépôts et consignations, déjà chargée du droit individuel à la formation des élus (Dife). Ce soutien financier pourrait être adossé au fonds de financement existant,

ne pouvions pas inscrire cette disposition dans le dur de la loi. C’est pourquoi nous demandons un rapport au Gouvernement en vue d’examiner l’opportunité d’un tel dispositif de réinsertion professionnelle et, au delà, d’évolution professionnelle. Il s’agirait tout simplement de compléter l’arsenal juridique permettant de sécuriser la sortie de mandat,

au moment de leur entrée dans le mandat, mais des élus qui, soit ayant évolué professionnellement, soit ayant mis entre parenthèses leur carrière professionnelle, souhaiteraient, à l’issue de leur mandat,

Madame la ministre, nous ne sommes pas vraiment d’accord avec

nous accepterons la vôtre, madame la ministre.

ou plutôt, devrais je dire, le non recours, à l’ADFM. En effet, comme je l’ai mis en évidence avec mes collègues Canayer et Lahellec dans notre rapport d’information relatif à la sortie de mandat des élus locaux, en dépit des efforts de publicité pour faire connaître cette aide,

Ces amendements, y compris donc le vôtre, visent à supprimer la prise en compte de la durée de suspension du contrat de travail dans l’ancienneté nécessaire pour certains droits sociaux. Je rappelle simplement en préambule que la période de la fin du mandat n’est pas forcément le moment le plus heureux dans la vie élective… Or la disposition

Aussi, à l’issue de ce dernier, retrouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations dans le cadre de leurs fonctions peut se révéler difficile. En conséquence, et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, nous proposons de réduire à un an la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

Une fois ce dernier achevé, il retrouve son précédent emploi et bénéficie notamment des avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat. Si le mandat est renouvelé, les dispositions relatives au retour à l’emploi précédent et à la récupération des avantages ne s’appliquent pas, sauf si la durée totale de la suspension a été inférieure à cinq ans. Ainsi, un salarié devenu député ou sénateur en début de mandature et qui est réélu pour la mandature suivante perd le bénéfice de ces dispositions, car il dépasse la durée totale de cinq ans de suspension. si un salarié devient député ou sénateur en cours de mandature, à la suite d’une démission, par exemple, il conservera le bénéfice de ces dispositions s’il est réélu pour la mandature suivante, mais dans la limite de cinq ans de suspension au total. Cependant, cette exception ne vise que les membres de l’Assemblée nationale, puisqu’elle se limite à cinq ans. Elle ne prend pas en compte, de fait, la durée d’un mandat de sénateur, qui est de six ans.

le salarié élu à l’Assemblée nationale ou au Sénat ayant au moins un an d’ancienneté à la date de son entrée en fonction peut obtenir la suspension de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat. Par ailleurs, aucun motif de refus n’est prévu par le code du travail. En d’autres termes, dès lors que le salarié satisfait la condition d’ancienneté d’un an, l’employeur ne peut s’opposer à cette suspension. À l’expiration de son mandat, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente. L’obligation de réemploi et le respect des avantages acquis ne sont pas exigés lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension du contrat ait été inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsqu’un salarié membre d’une assemblée parlementaire est élu dans l’autre. Le régime juridique

concrètement dans la planification écologique et de répondre à l’urgence sociale. Ce sont des femmes et des hommes qui sont sur le pont à 200 %, nous le savons tous, qui veulent faire vivre leur commune, animer leur département et aménager leur région. Madame la ministre, nous avons hâte de vous voir revenir

des attentes des élus locaux. Je veux le dire à l’ensemble des élus, et plus largement à toutes celles et à tous ceux qui s’interrogent ou qui vont s’interroger, dans les années qui viennent, sur la possibilité de se présenter aux élections, c’est un statut qui vise à protéger et à sécuriser.

sans tabou, de manière positive et forte. Maintenant, madame la ministre, nous vous confions ce texte. Si votre responsabilité est grande, notre attente l’est tout autant. Nous souhaitons que ce texte aille rapidement

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun. Mes chers collègues, en accord avec le Gouvernement,

quinze, la déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat et d’un vote sur cette déclaration, en application de l’article 50 1 de la Constitution, relative au débat sur l’accord de sécurité franco ukrainien et la situation en Ukraine. Y a t

– Kanaky, a demandé l’inscription, en second point de l’ordre du jour de son espace réservé du jeudi 21 mars, d’une proposition de résolution, en application de l’article 34 1 de la Constitution, invitant le Gouvernement à à reconnaître l’État palestinien et à agir pour un cessez le feu effectif et durable dans l’attente de négociations. Acte est donné de cette demande, qui sera inscrite à l’ordre du jour sous réserve de l’information préalable du Gouvernement. À la demande du groupe CRCE K, le temps de parole des groupes politiques pourrait être de 45 minutes. En outre, nous pourrions fixer le délai limite pour les inscriptions des orateurs des groupes dans la discussion générale au mercredi 20 mars à 15

Enfin, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande le retrait de l’ordre du jour du mardi 2 avril du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui en font la demande. Il demande également que la lecture des éventuelles conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative, ainsi que la nouvelle lecture du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, initialement prévues le 3 avril, soient inscrites en dernier point de l’ordre du jour du mardi 2 avril prochain. Le reste de l’ordre du jour préalablement fixé par la conférence des présidents lors de sa réunion du 14 février dernier est sans changement. Acte est donné de cette demande. En conséquence, s’agissant du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, le délai limite de dépôt des amendements serait fixé au mardi 2 avril prochain à 9 heures et le délai limite pour les inscriptions des orateurs des groupes au vendredi 29 mars,